La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 9 mai 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. avons terminé avec le débat sur les infrastructures routières à la suite de la présentation du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures du 1 février 2018. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur de la demande de débat dispose d'un temps de parole de huit minutes,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Républicains a souhaité l'inscription à l'ordre du jour d'un débat sur les infrastructures routières, à la lumière du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, pour rappeler son attachement à un réseau routier étendu, longtemps considéré comme exceptionnel, et qui continue à se développer.

Il est un atout formidable pour la mobilité dans nos territoires, à condition qu'il soit bien entretenu. Or nous le savons bien, mes chers collègues, une tendance à la dégradation du réseau routier national non concédé et du réseau autoroutier a été observée ces dernières années. Même si elle peut sembler limitée pour l'instant,

supérieure ou égale à 12 sur 20, ce taux a commencé à baisser en 2013, pour atteindre 84,5 %, puis 83,8 % en 2014 et 83,3 % en 2015. Cette dégradation de l'état du réseau routier a des conséquences sur le terrain, puisqu'elle se traduit par la multiplication des limitations temporaires de vitesse ou des mesures de restriction de la circulation.

consistent à réhabiliter, renforcer, renouveler ou reconstruire des ouvrages d'art et des chaussées de sections d'itinéraires fortement dégradées en raison de leur ancienneté ou d'événements climatiques. également à financer des opérations de mise en sécurité des tunnels routiers et le renouvellement des principaux équipements qui y contribuent, des aménagements de sécurité, des équipements dynamiques visant à améliorer la gestion du trafic par l'information des usagers et la régulation des accès des accès ou de la vitesse, ainsi que l'aménagement d'aires de service et de repos. Malheureusement, les précédents gouvernements ont eu tendance à promettre et même à engager la réalisation de nombreux projets d'infrastructures sans nécessairement s'assurer de leur faisabilité financière. Sur le plan budgétaire, cette politique s'est traduite par une inadéquation entre les ressources et les dépenses de l'AFITF. En effet, depuis 2013, l'AFITF rencontre des difficultés budgétaires. Celles-ci sont d'abord dues aux reports successifs de l'entrée en vigueur de l'écotaxe, puis à l'abandon de cette dernière, décidé à la fin de l'année 2014.

aucune recette supplémentaire. Les ressources de l'Agence ont ainsi fortement diminué, passant de 1,9 milliard d'euros en 2012 à 1,6 milliard d'euros en 2013 et 1,7 milliard d'euros Le manque à gagner résultant de l'abandon définitif de l'écotaxe n'a été que partiellement compensé par l'affectation d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE. Si cette fraction s'est élevée à 1,1 milliard d'euros en 2015, l'AFITF a dû assumer

En 2017, alors que les besoins de financement de l'Agence étaient estimés à 2,5 milliards d'euros par son ancien président, Philippe Duron, son budget s'est élevé à 2,2 milliards d'euros. est du réseau autoroutier, il revient aux sociétés concessionnaires d'entretenir le patrimoine qui leur a été confié et à l'État de vérifier que leurs obligations sont bien remplies. La qualité du réseau autoroutier est suivie grâce à des indicateurs que les concessionnaires d'autoroutes doivent renseigner depuis 2005 et que l'État contrôle au moyen de visites non formalisées, qui permettent de repérer des zones défaillantes, ainsi que d'audits approfondis. En ce qui concerne l'état du réseau, si la proportion des autoroutes en très bon état de surface est restée relativement stable- autour de 65 celle des autoroutes en bon état de surface a diminué depuis 2011, passant de 31 % à 18 % en 2013. En conséquence, la proportion du réseau autoroutier dont l'état est plus ou moins dégradé a augmenté, passant On observe donc une tendance à la dégradation d'une partie du réseau autoroutier, ce qui n'est pas acceptable. Dans son rapport sur les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes de juillet 2013, la Cour des comptes avait souligné l'expertise des services de l'État effectuent les contrôles relatifs à l'état du patrimoine autoroutier, tout en recommandant un renforcement de ces contrôles. Par ailleurs, elle avait relevé que l'État n'utilisait pas suffisamment les outils à sa disposition pour contraindre les sociétés concessionnaires à remplir leurs obligations. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite également replacer ce débat dans le cadre de l'aménagement du territoire. Nous le savons tous, un des préalables à tout renouveau des territoires est de les doter d'infrastructures modernes de communication, dont les routes et les autoroutes. Que seraient devenues la Bretagne, la Vendée, les vallées alpines, aujourd'hui prospères- pour ne citer que ces exemples emblématiques-, sans un investissement massif dans les infrastructures de communication, dont le financeur principal a été l'État ? Je suis un élu des Ardennes, territoire enclavé jusqu'en 2005, dépourvu d'investissements significatifs de la part de l'État en infrastructures de communication, sans doute parce que ce département était considéré comme la porte d'entrée des invasions à une époque où nos voisins n'étaient pas toujours nos amis,

! Pour mettre fin à cette situation pénalisante et remettre les Ardennes sur les grands axes de communication européens, le conseil général a dégagé d'importants crédits et a convaincu l'État et la région de l'aider à construire une liaison autoroutière qui permette d'arrimer

En plus de liaisons autoroutières, les territoires traversés doivent disposer des moyens de moderniser leurs réseaux routiers départementaux embranchés sur les échangeurs autoroutiers, afin que cet ensemble d'infrastructures permette d'atteindre l'un des objectifs en matière d'aménagement du territoire maintes fois rappelés par les spécialistes, à savoir qu'au moins 90 % de la population de notre pays doit avoir accès en moins de trente minutes à un échangeur autoroutier ou à une gare TGV. Pour conclure, je souhaite interroger le Gouvernement sur deux points essentiels qui touchent à la pérennité de nos infrastructures autoroutières et routières. Premièrement, qu'en est-il de la possible création d'un établissement public doté d'un financement issu du transport routier pour mener la rénovation du réseau national et la construction de nouvelles infrastructures routières et autoroutières ?

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'interviens aujourd'hui à nouveau devant votre Haute Assemblée pour poursuivre nos échanges autour des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, le COI. Le 13 mars dernier, j'avais déjà eu l'occasion de vous exposer les grands principes de la politique globale de mobilité que nous entendons promouvoir. Le 28 mars, nous avons pu débattre ensemble de l'avenir des lignes à grande vitesse et de l'aménagement du territoire. Vous me donnez aujourd'hui l'occasion d'aller plus loin en matière de politique routière, et je vous en remercie. Notre objectif est de bâtir une société de mobilité inclusive, dont chacun de nos territoires, chacun de nos concitoyens puisse tirer parti au quotidien. Faire face à ce défi, qui conjugue efficacité économique, aménagement du territoire et cohésion sociale, c'est naturellement donner à la route la place qui doit être la sienne la sienne au coeur d'une politique de lutte contre le changement climatique qui doit favoriser le développement des modes alternatifs pour le transport des biens et des personnes, des biens et des personnes, notamment le ferroviaire. Alors que 90 % du transport de marchandises et de voyageurs est à ce jour assuré par la route, le développement de ces modes alternatifs est une priorité fondamentale de la politique de mobilité que je Cela étant, n'oublions pas que le système routier français constitue un réseau de 1 million de kilomètres qui assure un maillage extrêmement fin de chacun de nos territoires. Par ailleurs, la route du XXI siècle n'aura que peu à voir avec celle qui a été cartographiée et développée par Daniel-Charles Trudaine au XVIII siècle. Demain, la route sera encore plus utile et pertinente, parce qu'elle sera plus propre, plus innovante, plus connectée et plus sûre. Elle devra favoriser le développement des véhicules électriques autonomes, du vélo, des nouveaux transports en commun à faibles émissions, du covoiturage, de l'autopartage et de la multimodalité. Lors de son discours du 1 juillet 2017 à Rennes, le Président de la République a fixé un cap très clair : recentrer nos politiques de mobilité sur les transports du quotidien, la lutte contre la congestion dans les grandes agglomérations, l'accès à l'emploi et aux services dans les territoires et l'organisation de nos systèmes logistiques. Comme vous le savez, les besoins de nos territoires, de nos concitoyens, de nos entreprises ont beaucoup évolué depuis vingt ans. Ils continuent à évoluer rapidement. Dans un contexte marqué par les contraintes qui pèsent sur les finances de l'État et des collectivités territoriales, la route du futur devra également être plus sobre. Nous devons anticiper et accompagner ces évolutions majeures en révisant en profondeur nos stratégies et nos modes d'action. Ce besoin de changement, votre Haute Assemblée l'appelle de ses voeux depuis longtemps. J'ai déjà eu l'occasion, à cette tribune, de saluer les travaux de votre commission des finances et de votre commission de l'aménagement du territoire

Cette impatience, je la comprends, je la partage, et je mesure l'urgence d'y apporter une réponse, afin d'éviter que ne se creusent les fractures sociale et territoriale. J'y insiste, la capacité de la route à devenir un facteur d'inclusion est l'un des grands défis de la mobilité de demain.

caractérisé depuis trop longtemps, il faut oser le dire, par les annonces et la fuite en avant, et par une technique bien connue en politique et bien éprouvée, qui veut que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ». C'est le sens du travail confié au Conseil d'orientation des infrastructures, présidé par Philippe Duron. Le rapport qui m'a été remis le 1 février dernier est le fruit d'un travail considérable. Je me réjouis que les conclusions issues de cette démarche exigeante aient été adoptées à l'unanimité des membres du COI et je salue ici l'engagement de vos collègues, Hervé Maurey, président de la Leur travail est d'autant plus précieux qu'il pose les bases d'une véritable stratégie d'investissement pour les deux décennies à venir. Comme vous le savez, trois scénarios sont désormais sur la table. Le premier, à ressources constantes, permet simplement de répondre aux besoins d'entretien du patrimoine existant. Le deuxième satisfait les priorités fixées par le Président de la République, mais au prix de moyens supplémentaires significatifs, à hauteur de 600 millions d'euros par an. Le troisième, enfin, prévoit une accélération des projets. il mobilise environ 80 milliards d'euros sur une période de vingt ans, soit un doublement des dépenses par rapport à la période 2012-2016 pendant au moins dix ans. Quel que soit le scénario retenu, le rapport recommande un certain nombre de priorités dans la façon de conduire nos politiques d'investissement. S'agissant des routes, le COI insiste à juste titre sur la priorité absolue que constituent l'entretien, la régénération du réseau routier national non concédé et la modernisation de son fonctionnement. Cette recommandation rejoint les conclusions de l'audit externe qui m'a été remis en avril 2018, lequel souligne l'état critique de ce réseau : 50 % des surfaces des chaussées sont à renouveler et près d'un pont sur dix est en mauvais état. Dans son rapport de mars 2017, le président Hervé Maurey tirait déjà la sonnette d'alarme en dénonçant « un réseau en danger ». Là encore, notre sous-investissement a été manifeste et, au rythme de l'effort actuel, deux décennies seraient nécessaires pour remettre en état l'ensemble du patrimoine. Qui pourrait s'en satisfaire ? Au-delà, l'enjeu de la modernisation de nos routes est également posé. Celle-ci doit favoriser le développement des véhicules connectés et autonomes et améliorer la gestion des flux de trafic. La première des priorités à laquelle je suis fondamentalement attachée est la desserte routière de nos territoires.

Il faut également avoir en tête que, si le réseau routier national supporte près d'un tiers des trafics, il ne représente que 2 % des infrastructures linéaires routières de notre pays. Sans chercher à se substituer aux collectivités locales, l'État doit leur apporter son soutien et poursuivre l'animation de la communauté routière pour développer et diffuser des techniques adaptées à des routes sobres, écologiques et peu coûteuses. Enfin, le COI nous invite à sortir de la logique du « tout ou rien », qui a longtemps prévalu dans la réalisation des grands projets. À nous désormais d'être innovants et raisonnables à la fois. Concevons et phasons intelligemment les projets pour les mener à bien et répondre efficacement aux problèmes de congestion en mobilisant les moyens compatibles avec nos finances publiques. L'équation n'est pas simple, mais elle n'a rien d'insoluble. Dans cette perspective, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures permet d'ouvrir une nouvelle page dans nos choix d'investissement, et ce afin de sortir des impasses financières et politiques sans renoncer à notre ambition collective en faveur de l'amélioration S'inspirant de ces recommandations, le Gouvernement fera très bientôt connaître ses choix. C'est notamment l'objet du futur projet de loi d'orientation sur les mobilités que je présenterai avant l'été. Ce texte proposera une stratégie d'ensemble, ainsi qu'une programmation sincère de nos infrastructures pour les deux prochaines décennies. Nous aurons l'occasion d'en reparler précisément lorsque votre Haute Assemblée sera invitée à examiner et à enrichir ce projet de loi. Dans le domaine routier, nous nous montrerons à la hauteur des défis qui sont les nôtres, si cette programmation sait conjuguer quelques objectifs aussi simples que fondamentaux.

Il faut en terminer avec les promesses non tenues, parce qu'intenables. Réhabiliter la parole publique passe par davantage de sincérité, en particulier en matière budgétaire. C'est raisonnable et possible. Je compte sur votre exigence pour nous accompagner dans cette louable entreprise, que j'aborde avec détermination et confiance. Mes chers

des chaussées, avec 40 % des surfaces à renouveler, et des ouvrages d'art, avec 30 % des ponts à réparer. En 2018, nous avons d'ores et déjà augmenté les crédits consacrés à l'entretien et la modernisation du réseau routier en les faisant passer à 800 millions d'euros, à comparer avec les 670 millions d'euros dépensés en moyenne au cours des dix dernières années. Toutefois, une action plus forte de remise à niveau est indispensable. Il nous faudra progressivement

et des équipements du réseau routier national non concédé. Ce plan devra être intégré à la future loi de programmation des infrastructures et devrait fixer des objectifs quantitatifs d'amélioration du réseau routier sur la base d'échéances quinquennales- 2022, 2022, 2027, 2032 et 2037-, ce qui permettra d'agir en faveur de la sécurité des usagers sur l'ensemble du réseau, mais aussi de travailler sur une massification et une industrialisation des chantiers. La parole

je vous remercie

en permanence. Enfin, le Val-d'Oise est un cul-de-sac pour la troisième grande structure à vocation circulaire qu'est la Francilienne pour l'Île-de-France. En effet, si la liaison vers l'est, à partir de Cergy en passant par Roissy, a été réalisée, sur l'initiative, d'ailleurs, du conseil départemental et avec le soutien financier de la région- cette époque est révolue-, le bouclage vers l'ouest, par le prolongement de Méry-sur-Oise jusqu'à Orgeval, dans les Yvelines, reste une ardente nécessité. À l'issue du débat public de 2006, l'État a retenu un tracé. Ce projet a été soutenu par l'assemblée départementale dans une motion unanime exprimant les attentes du département sur les communes d'Éragny et d'Herblay. Depuis l'avis de la commission Mobilité 21, le bouclage de l'A 104 a été classé dans les secondes priorités. Le rapport de Philippe Duron préconise de poursuivre les études de réalisation et de statuer à nouveau vers 2030 Cela s'apparente fort à un renvoi aux calendes grecques pour des raisons budgétaires qui n'échappent à personne. Madame la ministre, pensez-vous que la ville-monde que veut être le Grand Paris peut attendre 2050- en étant optimiste-pour disposer enfin du grand anneau périphérique de liaison entre les principaux pôles de la grande couronne parisienne et de contournement de la zone la plus dense ? Que deviendrait alors l'un des grands projets fondateurs du Grand Paris, le port Seine-Métropole Ouest, à Achères ? ? du développement du bassin de vie de la confluence Seine-Oise, d'ampleur comparable à l'agglomération rouennaise ? Enfin, quel est votre objectif en matière de programmation des étapes préalables nécessaires à la réalisation de cette grande infrastructure ? La la ministre. Monsieur le sénateur Bazin, je suis tout à fait consciente des enjeux liés à l'amélioration de la desserte du nord-ouest de l'Île-de-France. le projet de prolongement de la Francilienne entre Méry-sur-Oise et Orgeval soulève des difficultés importantes depuis de nombreuses années quant au choix du tracé et ses impacts environnementaux. Vous avez mentionné les contraintes budgétaires. Certes, il s'agit d'un projet estimé à 3 milliards d'euros, pour lequel aucun plan de financement crédible n'a pour l'instant été identifié. Mais, au-delà, si un certain consensus a pu se dégager dans le Val-d'Oise, le projet pose des difficultés importantes d'insertion dans les Yvelines. Comme vous le soulignez, depuis que la commission Mobilité 21 a classé ce projet en secondes priorités, quel que soit le scénario financier considéré, les études et la concertation n'ont pas été poursuivies. Le Conseil d'orientation des infrastructures a quant à lui mis en avant, outre les difficultés environnementales, la priorité à donner aujourd'hui aux solutions alternatives à la route dans le coeur de l'Île-de-France. Pour l'ensemble de ces raisons, et compte tenu des gains que l'on entend tirer de ce projet, il nous faut rechercher et privilégier l'optimisation du réseau existant et le report des usagers sur les transports collectifs, la réalisation du prolongement de l'autoroute

Madame la ministre, vous avez dit il y a quelques instants qu'il était temps de sortir de décennies de promesses non financées pour s'engager sur une trajectoire claire, cohérente et sincère qui réponde vraiment aux attentes des citoyens. Président de la région Guyane pendant dix-huit ans, je peux témoigner des paroles non tenues par les gouvernements successifs qui se sont engagés à désenclaver le territoire par la route du fleuve reliant le littoral à Maripasoula. Dans cette commune

kilomètres restent aujourd'hui à construire et figurent à ce titre dans le schéma d'aménagement régional validé par le Conseil d'État. Dans son rapport, le Conseil d'orientation des infrastructures juge prioritaire de réduire les inégalités territoriales en prenant en compte les besoins spécifiques des outre-mer, notamment à travers les assises de l'aérien et celles des outre-mer. Vous le savez, les caractéristiques géographiques, climatiques et démographiques de nos territoires ne sont pas sans incidence sur la construction et l'entretien des réseaux routiers se révélant très coûteux. et sans présager du résultat des Assises, j'aurais aimé avoir votre sentiment, madame la ministre, sur le développement des infrastructures routières en vue du désenclavement des outre-mer, en particulier en Guyane. Cette problématique aura-t-elle toute sa place dans le projet de loi d'orientation sur les mobilités ? Si nous devons naturellement avoir recours au transport aérien et au transport fluvial, je reste convaincu que le véritable désenclavement, celui qui participe activement au développement économique et social d'un territoire, passe nécessairement par la route.

Celles-ci sont l'occasion de mettre en lumière les enjeux majeurs que représentent l'accessibilité et le désenclavement pour les territoires d'outre-mer. Je suis personnellement très attachée à ces questions. En ce qui concerne la Guyane, le plan d'urgence mis en place en 2017

Les services de l'État en Guyane sont également pleinement mobilisés pour faire avancer les études et les procédures qui permettront, à terme, l'aménagement à deux fois deux voies de la RN 1 et de la RN 2 à la sortie de Cayenne, aujourd'hui soumises à des congestions très importantes. Comme vous pouvez le constater, nous partageons avec vous l'ensemble de ces enjeux et l'État est au rendez-vous de ses engagements. La parole

actionnaires des autoroutes ? Timidement, le rapport Duron indique que l'anticipation de la fin des principales concessions autoroutières mérite d'être examinée dès à présent cela doit même constituer une priorité absolue. Si la politique des transports a souffert des promesses non financées, elle a peut-être surtout souffert de cadeaux faits au privé, comme s'apprête encore à en à travers le nouveau pacte ferroviaire. Il suffirait aujourd'hui de dénoncer ces concessions et d'indemniser les concessionnaires pour reprendre la main sur un rendement de 1 à 2 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas une bagatelle. Nous avons déposé une

Pour autant, les contrats des sociétés concessionnaires ont été modifiés pour y insérer des clauses plafonnant la rentabilité desdites sociétés qui peuvent conduire à réduire la durée des concessions ou à limiter- voire à baisser-les tarifs de péage. Des indicateurs de performance ont également été introduits dans les contrats. Par ailleurs, depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité

lesquels des parlementaires, le président du conseil départemental et la représentante de la région Occitanie, afin de vous convaincre de la nécessité de porter à deux fois deux voies la RN 88 reliant Toulouse à Lyon.

de circulation sécurisées et confortables, avec des temps de parcours fiables. Comme vous l'avez rappelé, nous avons eu l'occasion d'en discuter au mois de mars dernier avec le président du conseil départemental de l'Aveyron.

madame la ministre, mes chers collègues, l'une des priorités figurant dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures porte sur le développement de la performance des transports et la lutte contre la congestion routière et la pollution. En accord avec cette proposition, je souhaite attirer votre attention, madame la ministre, sur le problème national de la congestion numérique des infrastructures routières. En effet, l'utilisation massive des technologies d'information du trafic en temps réel

visant le trajet le plus court et/ou le moins cher. Cette situation provoque des dégradations irrémédiables pour les voiries locales. Les collectivités, dans le contexte budgétaire que nous connaissons, peinent à faire face à ce phénomène. Les riverains sont bien sûr affectés de plein fouet par ces reports numériques du trafic : bruit, insécurité, pollution de l'air, dépréciation de l'immobilier ... Par ailleurs, la recrudescence des véhicules utilitaires légers sur nos routes, liée à l'explosion de la vente par internet, renforce ce surplus de trafic. Et c'est sans compter le coût environnemental induit ! L'efficacité du transport routier de marchandises ne peut se faire au prix d'une aggravation des conditions de vie de nos concitoyens et au mépris des infrastructures financées par les collectivités. Les élus locaux tentent bien de couper le trafic à coup d'arrêtés d'interdiction de circulation. Mais cela ne fait qu'entraîner de nouveaux reports et ne règle pas le problème à la racine. Afin de conserver un niveau satisfaisant de service et de ne pas accroître

Ce dispositif a été conçu de manière concertée avec les opérateurs privés. Les échanges se poursuivent pour améliorer la qualité de l'information routière.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les besoins en matière d'entretien des routes françaises sont bien connus et le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures appelle à financer l'innovation routière pour ne pas être dépassé. L'état du réseau routier est aujourd'hui encore très convenable. Toutefois, plusieurs rapports ont souligné la baisse des dépenses consacrées à la voirie par les collectivités : de 2013 à 2015, elles ont chuté de 19 %, soit 15 milliards d'euros, en partie en raison d'une baisse des dotations Cette somme représente à peine 0,6 % de la valeur totale du patrimoine routier national. À ce rythme, il faudrait donc cent soixante années pour renouveler l'ensemble du réseau. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation : priorité devra donc être donnée aux transports du quotidien. L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs va redessiner la carte de France des mobilités locales. Le rapport préconise en conséquence de miser sur quelques lignes à haute performance. Mais c'est oublier que la France, c'est aussi un tissu territorial de 36 000 communes qui communiquent entre elles. La promotion de ces axes routiers et le déploiement d'une nouvelle palette de routes locales sont donc complémentaires pour assurer la vitalité de nos territoires. Madame la ministre, la prochaine ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs va appauvrir la desserte de certains territoires. Les grandes lignes seront sauvées et le Gouvernement s'est engagé à assurer le maintien des petites lignes. Cette promesse pourra-t-elle être tenue ?

Or, lors de la récente inauguration de la liaison entre l'A 6 et l'A 89, Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur, a indiqué que le contournement ouest de la ville de Lyon, qu'il avait pourtant lui-même défendu, contournement reliant l'A 6, au nord, à l'A 7, au sud, ne se réaliserait finalement jamais. On connaît pourtant tous les méfaits de l'étranglement du fameux tunnel de Fourvière, qui fait de Lyon une grande capitale du bouchon ! Il semble que ce soit maintenant exclusivement par l'est que s'esquisse progressivement un grand contournement un grand contournement routier de l'agglomération lyonnaise, lequel engendrera- mais je devrais dire « amplifiera » -des conséquences lourdes pour le département de l'Ain au regard des reports de circulation qui vont s'opérer et des nuisances associées.

la métropole lyonnaise souhaite pouvoir réduire le trafic traversant le coeur de son agglomération et le déplacer sur un autre itinéraire, afin de transformer l'axe A 6-A 7 en boulevard urbain. Les premiers résultats des études privilégient l'hypothèse d'un contournement par l'est, qui mobiliserait moins de crédits à court terme et qui pourrait être lancé plus rapidement. Ce contournement comporterait des aménagements sur les réseaux concédés d'une valeur comprise entre 260 et 680 millions d'euros dont la faisabilité doit encore être confirmée.

Les élus des territoires concernés ont participé à une réunion organisée le 23 février dernier. Je veillerai à ce qu'il en soit de même lors des futures réunions sur le projet. Dans ce cadre, il sera utile de disposer d'une véritable comparaison de l'ensemble des éléments sur toutes les solutions. dans la concertation, et en liaison étroite avec les acteurs locaux, arrêter une stratégie de long terme sur ces trafics de transit autour du noeud lyonnais.

à aborder des questions, certes importantes pour nos territoires, mais de nature très différente des sujets nationaux qui concentrent votre attention. L'autoroute Castres-Toulouse a fait l'objet d'un engagement depuis plusieurs années.

des territoires de l'est toulousain. Il s'agit vraiment d'un très bel exemple de ce que doit être notre politique en termes de mobilité. Je me rends à Toulouse jeudi. J'aurai l'occasion de vous y rencontrer avec les membres du conseil régional et les présidents des conseils départementaux,

adaptée aux besoins de la population et de l'économie locale, et favoriser ainsi une meilleure structuration de l'aire métropolitaine toulousaine, en soutenant le développement d'un réseau de villes moyennes organisé en étoile autour de Toulouse. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a été menée au début de

680 a été signé le 22 décembre 2017. S'agissant de la section Verfeil-Castres, un important travail d'étude et de concertation avec les acteurs locaux était nécessaire pour lever les réserves formulées

par des partenariats public-privé, qui prennent la forme de concessions ou, plus rarement, de marchés de partenariat. Dans ces deux cas, l'État confie à un partenaire privé une mission globale. Pour une concession, les recettes proviennent du paiement des péages par les usagers. Pour un marché de partenariat, la rémunération du partenaire privé est assurée par un loyer financé par le contribuable. En dix ans, les tarifs des péages ont connu une hausse de plus de 20 une augmentation supérieure à l'inflation. Le 1 février dernier, ces tarifs ont encore augmenté de 1 % à 4 %. Ces augmentations sont difficilement acceptables lorsque l'on sait que, dans le même temps, les sociétés privées autoroutières se portent particulièrement bien, avec une rentabilité élevée qui se situe entre 20 % et 24 %. L'ARAFER avait d'ailleurs indiqué que les augmentations des tarifs de péages prévues excédaient le juste niveau qu'il était légitime de faire supporter aux usagers. estimait notamment que le niveau de rémunération des sociétés concessionnaires devait être plus conforme aux risques supportés. À titre d'exemple, le coût du trajet sur l'A 28 entre Rouen et Alençon coûte 23,70 euros pour 161 kilomètres. Le nouveau plan d'investissement autoroutier devrait être l'occasion d'amender certaines clauses du cahier des charges des conventions de concession. Madame la ministre, vous venez de réaffirmer le rôle régulateur de l'État, qui imposerait des critères

ce débat sur les infrastructures routières, à la suite de la présentation du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, était plus que nécessaire tant ses conclusions ont été arrêtées arbitrairement, sans aucune concertation préalable avec les élus locaux. Comme en 2012 et la fameuse commission Mobilité 21, l'État revient sur ses engagements en supprimant des opérations pour lesquelles il avait pourtant contractualisé un financement avec les collectivités locales.

Rien que ça ! Ainsi, cette liaison autoroutière, dont le principe a été arrêté en 1987, afin de relier l'A 7 et l'A 9 par le sud d'Avignon, resterait en l'état.

Autant vous dire, madame la ministre, que la réaction de tous les élus concernés a été violente, solidaire et déterminée. Les députés d'Avignon et de Châteaurenard ont d'abord rencontré votre directeur de cabinet, M. Papinutti. Puis, le 14 mars dernier, une imposante délégation composée du maire d'Avignon, du président de l'agglomération, des cinq parlementaires locaux, ainsi que des représentants des deux départements et de la région s'est rendue à Matignon pour saisir le Premier ministre de ce dossier.

Les projets qui se déroulent dans le cadre des contrats de plan ont vocation à être poursuivis dans ce cadre. Je suis bien consciente de l'importance des problèmes de congestion

Roumazières-Loubert-Exideuil-sur-Vienne, avec la réalisation de la première phase d'ici à 2020, et de préparer la réalisation de la seconde phase entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Roumazières-Loubert, en effectuant les études et acquisitions foncières, ainsi que les travaux préparatoires. On s'en souvient, le 20 septembre dernier, vous annonciez une augmentation de 100 millions d'euros de l'enveloppe des crédits de l'État affectés en 2018 à l'entretien des routes, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à 2017. Madame la ministre, ma question est la suivante à la fois de cette annonce d'une augmentation considérable des crédits de l'État alloués au domaine routier et de l'état catastrophique de la ligne ferroviaire entre Angoulême et Limoges- je vous rappelle que les trains ne circulent plus sur cette ligne depuis plusieurs semaines-, peut-on espérer que les aménagements de l'axe routier Angoulême-Limoges, qui est aussi l'axe reliant Limoges à la capitale bordelaise, puissent bénéficier de moyens financiers supplémentaires de la part de l'État ? Peut-on également espérer une avancée plus rapide des travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la RN 141, notamment pour la réalisation

en matière de fiabilisation des temps de parcours, d'amélioration de la sécurité routière et de la qualité de vie des riverains. La RN 141 correspond à la section ouest de la route Centre Europe Atlantique, qui est une liaison transversale très importante pour le réseau national français, rattache la façade atlantique au sillon rhodanien. Compte tenu des niveaux de trafic supportés et des enjeux que je viens de rappeler, cet axe a clairement vocation à être progressivement aménagé en deux fois deux voies. Cet aménagement Cet aménagement est aujourd'hui bien avancé, puisqu'il est réalisé aux trois quarts sur l'itinéraire entre Royan et Limoges. Il se poursuit grâce à la mobilisation de plus de 150 millions d'euros

S'agissant de la section La Vigerie-Villesèche, les travaux ont démarré à l'automne 2016, avec la construction d'un ouvrage d'art, et se poursuivront en 2018. Pour ce qui concerne la section Chasseneuille-sur-Bonnieure-Exideuil-sur-Vienne,

sur la RN 135. Vous me direz que c'est un petit bout de route nationale entre la RN 4 et la coquette préfecture de la Meuse, Bar-le-Duc, et que je ne fais

Ce projet de RN 135, qui connaît une évolution lente depuis une vingtaine d'années, mais certes comparable au rythme de toutes les réalisations nationales en la matière, doit

ne pas reporter à 2021 le début effectif des travaux. Deuxièmement, il faut intégrer cette réflexion dans une réflexion d'ensemble sur la desserte du site de Cigéo. La parole est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur Gérard Longuet, vous m'interrogez sur les intentions du Gouvernement concernant la RN 135. En effet, cette route nationale fait partie des mesures d'accompagnement du projet Cigéo.

à Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois. L'État a anticipé l'augmentation du trafic liée au développement du secteur de Bar-le-Duc et a déjà réalisé le contournement de la ville et la déviation de Longeville-en-Barrois. L'autre extrémité du barreau, au droit de Ligny-en-Barrois, sera également traitée avec la mise en oeuvre de la déviation de Velaines, actuellement inscrite au contrat de plan pour un montant de 48 millions d'euros, dont un peu plus de 27 millions d'euros de l'État. Une convention de financement vient d'être signée entre l'État et les collectivités. Cette opération doit se poursuivre avec des travaux préparatoires qui pourraient débuter en 2019. Il nous faut encore examiner, en lien avec le projet Cigéo, les aménagements qui pourront être réalisés sur les morceaux manquants, la déviation de Tronville-en-Barrois et l'aménagement à deux fois deux voies entre Longeville-en-Barrois et Tannois. Nous devrons disposer

le projet de création de l'autoroute A 831 pour relier la Vendée et la Charente-Maritime a été abandonné par Ségolène Royal, dont vous étiez la directrice de cabinet à l'époque. Ce projet prévoyait la création d'une autoroute de 64 kilomètres entre Fontenay-le-Comte et Rochefort, afin de désengorger les routes entre la Vendée et la Charente-Maritime, notamment pendant la période estivale. L'État s'était engagé à soutenir une alternative à cette autoroute. À ce jour, et malgré de nombreux échanges avec les collectivités locales, aucune hypothèse, notamment sur le volet financier, ne recueille l'assentiment des parties. Au regard de l'abandon de ces différents projets pour le Grand Ouest, je souhaiterais tout d'abord connaître les pistes de réflexion sur lesquelles le Gouvernement travaille, afin de proposer une offre de mobilité adaptée à nos territoires et à leur attractivité touristique.

pour une collectivité locale, de concéder l'une de ses infrastructures routières dans le cadre d'un projet de développement ou de modernisation lourde. En effet, cette possibilité n'est actuellement pas ouverte dans la loi. Le COI considère que la mise en oeuvre d'une telle proposition serait un moyen pertinent de portage pour certains projets.

Ces scénarios s'appuient sur le réaménagement du réseau départemental existant. Un protocole avait été préparé sur cette base, mais nous n'avons pas reçu l'aval des élus, qui s'interrogeaient sur le niveau de participation de l'État et souhaitaient conserver un projet de mise à deux fois deux voies sous statut autoroutier. Pour autant, je vous confirme que le projet d'amélioration de la desserte de ce territoire n'est pas abandonné. Le Gouvernement est naturellement prêt à rouvrir les discussions avec les élus pour trouver un aménagement permettant de faciliter les déplacements entre Nantes et La Rochelle, en complément de la

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le maillage routier est un levier d'attractivité important pour nos territoires, notamment pour ceux qui sont situés en zone rurale.

l'ancien ministre Jean-Pierre Soisson, à savoir la liaison Bourges-Auxerre-Troyes, qui a été abandonnée, ou au projet de liaison entre Bourges, Châteauroux et Poitiers

en précisant que « le réseau routier n'a pas évolué ces dernières années ». Lors de son audition au Sénat, M. Duron a insisté sur le fait que les infrastructures devaient être phasées, car le temps n'était plus aux promesses, mais à la mise en oeuvre.

Nos routes constituent aussi un patrimoine national. Et ce patrimoine national, comme tout patrimoine, doit être entretenu. Hélas, on peut remarquer, çà et là, qu'il est moins entretenu qu'avant.

prononcer, tout en vous souhaitant, madame la ministre, de pouvoir trouver des fonds pour tenir vos promesses avant 2025 !

La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, samedi notre pays a été frappé par un nouvel acte de barbarie de l'islamisme radical, au coeur de Paris. Le bilan, encore une fois, est lourd : une personne est décédée, quatre autres ont été blessées.

je souhaite une fois de plus rendre hommage et exprimer notre gratitude à nos forces de sécurité, qui ont neutralisé très rapidement le terroriste. Ce nouvel attentat nous rappelle le haut degré de menace qui continue de peser sur notre pays. Face à cette menace et à l'heure où la violence se déchaîne à travers le monde, comme nous l'avons encore constaté ces jours derniers, je veux dire, au nom du Sénat tout entier, que nous ferons face, que nous resterons unis et déterminés à poursuivre le combat et à défendre nos valeurs. Il y a un instant, dans le jardin du Sénat, je rendais hommage aux étudiants et aux lycéens qui se dressèrent contre le totalitarisme le 11 novembre 1940. Je pense, en cet instant, à nos soldats, à nos forces de sécurité, qui sont aux avant-postes de la liberté. Ce sont les mêmes valeurs qui nous rassemblent. Monsieur le Premier ministre,

et unis face à cette menace qui ne baisse pas d'intensité et qui ne baissera pas d'intensité dans les semaines et les mois à venir. Je vous invite à observer un moment de recueillement en hommage aux victimes de cet attentat.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, il y a soixante-dix ans, David Ben Gourion proclamait la création de l'État d'Israël. Pour celles et ceux qui avaient entendu Theodor Herzl théoriser l'« État des Juifs », cinquante ans auparavant, pour celles et ceux, peu nombreux, qui avaient échappé à la Shoah, ce fut ce jour-là un immense espoir, une délivrance et un accomplissement. Nous aurions aimé retrouver cette atmosphère. Au lieu de cela, depuis hier, nous avons en mémoire des images difficiles de morts par dizaines et de blessés par milliers, au moment même où était inaugurée à Jérusalem l'ambassade des États-Unis. Ces images succèdent à celles d'échanges de tirs de missiles et de contremissiles dans le ciel syrien, visant des cibles iraniennes ou des avions de Tsahal. Après avoir reçu Benyamin Netanyahou en décembre dernier et le prince héritier saoudien il y a un mois, le Président de la République a rencontré Donald Trump, président des États-Unis, voilà quinze jours. Le Président de la République a sans nul doute cherché à convaincre, à faire partager les préoccupations de la France. Il a sûrement été écouté, mais il n'a pas été entendu.

des mineurs, et près de 2 700 blessés, dont beaucoup par balles. La France condamne évidemment et sans aucune ambiguïté ces violences. si nous sommes sans aucune ambiguïté attachés à la sécurité d'Israël, nous ne pouvons pas accepter un tel niveau de violence face au droit fondamental des Palestiniens à manifester pacifiquement. La politique de la France est connue ; elle est ancienne. Elle a pour objectif la coexistence de deux États, Israël et la Palestine, vivant dans la paix et dans la sécurité au sein de frontières reconnues, avec Jérusalem pour capitale commune.

et multiplié les contacts avec le roi de Jordanie, avec le président Abbas et, aujourd'hui, avec le Premier ministre israélien.

considérons que cette décision n'apporte rien à la recherche de la solution durable que j'évoquais à l'instant. Dans cette région

Nous sommes au bord du gouffre. Il est urgent d'éviter une nouvelle escalade et d'établir enfin une paix durable. En effet, dans cette région déjà soumise à de fortes tensions, il y a tout à craindre d'une radicalisation et et d'une contagion du conflit. Nous le savons, la France est très engagée dans la recherche d'une solution politique et elle soutient la cause du peuple palestinien, dont les aspirations sont légitimes, mais aussi le droit d'Israël à la sécurité.

Il a appelé tous les responsables à la modération et à l'apaisement et a insisté sur la nécessité que les manifestations des prochains jours demeurent pacifiques. Au-delà, lorsque la sérénité sera revenue, comme nous l'espérons, il faudra redonner vie au processus de paix, car il n'y a pas d'autre solution durable que celle d'une paix juste et négociée entre deux États, garantissant une quiétude mutuelle à la Palestine et à Israël.

Jean-Yves Le Drian, qui est en route pour Bruxelles, où se tient une réunion importante avec M. Zarif, le ministre des affaires étrangères iranien, et nos partenaires européens signataires de l'accord de Vienne.

et Social Européen. Ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Madame la ministre, vous avez réuni hier les représentants des médecins urgentistes pour lancer une concertation sur les moyens

Sur les réseaux sociaux, des témoignages relatent des expériences malheureuses avec les services du SAMU. Pour autant, il importe de ne pas généraliser et de rappeler que, dans l'immense majorité des cas, les appels conduisent à une prise en charge rapide et efficace, dans le respect du patient. Les assistants de régulation et les médecins urgentistes font un travail difficile. Sous tension, ils traitent jusqu'à 700 appels par jour. C'est justement parce qu'il s'agit d'une mission primordiale, avec un nombre d'appels en augmentation auxquels il faut apporter une réponse humanisée, tout cela dans le respect d'une légitime exigence de sécurité, qu'il nous appartient de moderniser ce service pour tendre vers une prise en charge homogène et optimale pour les patients et en toute sécurité pour les professionnels.

Trop souvent, les assistants de régulation médicale se retrouvent en première ligne sans formation ni expérience suffisantes. Ensuite, la création d'un numéro unique pour toutes les urgences a été évoquée. Cela permettrait une meilleure lisibilité pour les patients et une plus grande efficience des services, en réduisant le délai entre l'appel et l'intervention. Enfin, même si elle est complexe- je sais que le Gouvernement peine pour l'instant à trouver des réponses-, la question de l'optimisation des moyens doit être abordée

La révolte du peuple de Palestine- des pierres contre des armes-est justifiée au regard de toutes les provocations de l'État israélien, provocations alimentées par les États-Unis, avec l'installation de leur ambassade à Jérusalem.

Vous avez su dénoncer le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem dans cet hémicycle. C'est très bien, mais il est temps maintenant d'agir fermement contre les exactions de l'État d'Israël. Il faut aujourd'hui faire cesser le massacre des jeunes Palestiniens, les placer sous protection de l'ONU, abroger le blocus de Gaza et reconnaître enfin l'État palestinien

Ce rapport montre une évolution récente, toujours plus marquée, vers l'augmentation des dividendes au détriment des salaires, mais aussi des fonds propres, voire du financement des investissements dans les grands groupes cotés. Cela doit nous interpeller collectivement. Nous avions, par le passé, essayé de revenir pour partie sur cet état des choses, notamment en faisant en sorte de rapprocher la fiscalité française sur les dividendes de celle qui s'applique aux revenus salariaux.

Vous deviez « libérer et protéger ». Pour ce qui est de libéraliser l'économie, nous avons vu ! Protéger les salariés, protéger la capacité d'investissement et les fonds propres des entreprises, et même protéger, en un sens, l'économie de marché contre elle-même, voilà les objectifs que vous pourriez vous fixer à l'avenir, monsieur le ministre

pour promouvoir le modèle rhénan de l'entreprise allemande-on nous parle souvent de l'Allemagne ! -, qui privilégie le long terme plutôt que le retour immédiat sur investissement, et donner ainsi enfin un contenu concret à ce qui n'est aujourd'hui qu'un concept : la protection des salariés ? La parole

qui réclament un niveau de rémunération plus élevé. Pour notre part, nous mettons en place une fiscalité attractive pour développer un actionnariat national indépendant, pour développer l'actionnariat salarié dans les PME,

Mardi dernier, Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Immédiatement, le département du Trésor a annoncé le rétablissement, sous trois sanctions économiques contre toutes les entreprises qui travailleraient avec l'Iran. En application du droit américain, toute entreprise, américaine ou non, qui passera outre ne pourra plus exercer ses activités aux États-Unis et sera sanctionnée de manière prohibitive.

Nos entreprises payent déjà depuis trop longtemps le prix de l'extraterritorialité du droit américain. Je pense bien sûr à l'amende de 9 milliards de dollars acquittée en 2014 par la BNP, ainsi qu'aux affaires Alstom, Total, Crédit Agricole, et j'en passe passe ... Depuis 2008, les entreprises européennes ont payé plus de 20 milliards de dollars d'amendes à la justice américaine ! Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement nos grands groupes, comme Airbus, Renault ou Accor, qui sont menacés qui sont menacés : nos PME et nos entreprises de taille intermédiaire font également l'objet d'un chantage économique inacceptable ! Benjamin Constant disait qu'il vaut mieux souffrir de l'oppression de ses ennemis que rougir des excès de ses alliés. Les États-Unis sont nos alliés, nos amis même, depuis leur naissance. Mais cela ne veut pas dire que nous devons tout accepter, au contraire

Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison : les sanctions extraterritoriales américaines sont inacceptables. Elles sont contraires au principe de liberté du commerce,

J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le secrétaire au Trésor américain pour lui demander des exemptions, des délais supplémentaires, ainsi que le respect des contrats conclus de bonne foi, dans le cadre de l'accord signé avec l'Iran, par les entreprises françaises implantées dans ce pays.

indépendante lui permettant de faire librement du commerce où elle le veut, quand elle le veut, sans dépendre des institutions financières américaines enfin,

L'horreur se répète : un attentat de plus, qui a donné lieu à de grandes et belles phrases. Un philosophe a parlé de « sidération rituelle ». La consternation et les indignations légitimes ne sont plus suffisantes. On a le sentiment que l'accoutumance au terrorisme islamiste nous guette. Or il y a pire que l'horreur : l'accoutumance à l'horreur ! Les réponses au terrorisme sont, bien sûr, techniques. La qualité du travail des forces de l'ordre et des services de renseignement mérite d'être saluée. une véritable réponse passe aussi, et surtout, par un réarmement moral et culturel de notre pays. Elle passe par la désignation claire et sans ambiguïté des causes et des racines du mal. Nous ne gagnerons la guerre contre l'État islamique, contre l'islam radical, contre l'islam politique, que si nous avons la volonté et le courage d'imposer partout et toujours nos valeurs républicaines Nous ne réglerons pas la question des attentats si nous laissons des quartiers entiers de notre territoire échapper aux lois de la République. L'urgence est de lutter avec une fermeté sans faille contre une certaine police de la pensée qui entrave notre liberté et conduit certains esprits vers l'islam radical.

immédiate de nos policiers, qui sont intervenus en moins de neuf minutes, nous aurions

Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas, dans nos grandes villes, à la fois des quartiers prospères et des quartiers qui se paupérisent, se ghettoïsent ; en effet, à force de vivre côte à côte,

Elle concerne la mortalité catastrophique qui touche en ce moment les abeilles. Voilà dix jours, j'étais avec les apiculteurs bretons, à Rennes, pour assister à l'arrivée d'un « convoi mortuaire », organisé pour alerter sur les pertes massives de colonies.

Sachant que la perte moyenne, pour chaque ruche, s'élève à 400 euros, je vous laisse imaginer la détresse, à la fois économique et humaine, de nos apiculteurs. Monsieur le ministre, ma question est double. Un plan d'urgence va-t-il être mis en oeuvre pour soutenir les apiculteurs, compenser les pertes de marge brute et aider à reconstituer les cheptels ? cheptels ? Sur un plan plus structurel, les causes de cette mortalité sont connues : elles sont en grande partie liées à notre modèle agricole intensif, fondé sur l'agrochimie.

dégradée dans leurs ruchers en sortie d'hiver. Les mécanismes de surveillance dont disposent actuellement les pouvoirs publics ne permettent pas de corroborer une généralisation de cette dégradation.

un observatoire des mortalités et des affaiblissements de l'abeille mellifère, ou OMAA. L'objectif est de mieux prendre en compte la situation sanitaire et d'identifier les facteurs de risque. Tous les apiculteurs bretons ayant constaté des mortalités ou des affaiblissements dans leurs ruchers sont invités à les déclarer au guichet unique qui a été mis en place. déclaration déclenchera une visite vétérinaire. Les résultats de la première année de fonctionnement de cet observatoire seront présentés au cours du dernier trimestre de 2018.

alimente le dispositif de pharmacovigilance animé par l'ANSES. Le 25 avril dernier, le Gouvernement a présenté son plan d'action sur les produits phytopharmaceutiques concernant les pollinisateurs. Sur la base d'un avis de l'ANSES, qui sera saisie prochainement, il est prévu de renforcer les dispositions relatives aux conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, en vue de protéger les abeilles domestiques et les insectes pollinisateurs. C'est mal

L'interruption du trafic deux jours sur cinq entrave également l'activité de la journée suivante. Le potentiel de nuisances de la grève pour nos entreprises est inacceptable. Les industries seront touchées à hauteur de près de 60 %. La France perd des marchés, faute de pouvoir les honorer.

de ce secteur de recourir à des modes de transport alternatifs, routiers et fluviaux, dont on voit bien les limites en termes d'augmentation de la durée d'acheminement et de surcoût financier- entre 5 et 20 euros par tonne. Le pire est à venir : les entreprises sont contraintes de puiser dans leurs stocks et, faute de pouvoir être transportées, les récoltes de juillet vont engorger des silos déjà saturés. Des mesures d'urgence s'imposent. Je vous demande de mettre en place un service minimum de fret ferroviaire en cas de grève pour toutes les industries, ... Ben voyons ! ... de prioriser les flux agricoles, de mettre en place des moyens importants pour moderniser les infrastructures fluviales et de prendre une mesure immédiate d'autorisation exceptionnelle de la circulation des camions les dimanches et jours fériés, à partir de vingt-deux

environ un tiers des trains de fret circulent. Pour le fret, deux jours de grève, c'est une semaine d'activité de perdue. L'État et SNCF Réseau sont pleinement mobilisés. Un guichet unique pour les entreprises J'ai par ailleurs demandé aux préfets d'être particulièrement vigilants, de signaler toutes les situations critiques pour les activités économiques et d'accorder, comme vous le préconisez, des dérogations pour la circulation des poids lourds le dimanche si

par décret du 27 juin 2017, vous proposiez un élargissement du champ des dérogations à l'organisation de la semaine dans les écoles maternelles et primaires permettant au directeur académique, sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou de plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine sur quatre jours.

des charges budgétaires qu'ils n'avaient pas prévues au regard des décisions d'un ou de plusieurs conseils d'école, mais surtout d'une baisse des dotations de l'État qui est aujourd'hui une évidence et que nous ne cesserons de rappeler ! Mes questions, monsieur le ministre, sont simples. Dès lors qu'un décideur-payeur n'aura pas été écouté, comment l'État assumera-t-il la charge créée de son seul fait ? Comment comptez-vous demander à vos services de se mobiliser pour permettre à ces territoires, aujourd'hui à deux vitesses, de retrouver une cohérence éducative territoriale ? Pourquoi n'avez-vous pas envisagé d'associer aux commissions prenant ces décisions les élus, qui sont, je le rappelle, les principaux payeurs, mais également les porte-parole, en matière de cohérence éducative, d'un territoire qu'ils connaissent et que ne représente pas toujours le conseil d'école ?

Lors d'une récente intervention télévisée, à l'occasion de sa visite à Berd'huis, le Président de la République a déclaré que, en 2018, le montant des dotations attribuées aux collectivités ne subirait pas de baisse, et connaîtrait même une augmentation, légère il est vrai.

À ce stade, aucune explication n'a été fournie et le constat est fait que, au plus haut des services de l'État, on ne communique pas les éléments qui permettraient de comprendre le mécanisme d'évolution des dotations en jeu. : le ministre de l'intérieur est-il déterminé à faire en sorte que la plus grande clarté soit faite et que les éléments de compréhension et d'analyse de ces évolutions des dotations soient rendus accessibles aux élus et à leurs associations ? Quelles corrections sont envisageables afin d'empêcher les redistributions sans cause réelle auxquelles on assiste et de rétablir une DSR plus équitable ? Quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet ? Il y va de la crédibilité de la parole de l'État. La parole

Elle est répartie en fonction d'un certain nombre de critères. Elle est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel fiscal par habitant inférieur

Madame la ministre, le dimanche 29 avril, le département de l'Aube a été frappé par une tempête de forte intensité. Plusieurs communes ont été impactées et les dégâts sont considérables. Plus de 140 maisons et quatre sociétés ont été touchées, sans parler des dommages paysagers et matériels. Une entreprise est complètement détruite, ce qui laisse une soixantaine de personnes au chômage technique. La loi du 13 juillet 1982 dispose que les personnes physiques ou morales victimes de catastrophes naturelles peuvent être dédommagées par leur société d'assurance pour les dégâts subis. Les communes les plus sinistrées ont ainsi envoyé à la préfecture une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Comment défendre les demandes des élus concernés quand aucun relevé de vitesse de vent n'a été réalisé aux endroits les plus touchés, sachant qu'il peut y avoir des pointes à 215 kilomètres-heure au centre de la tornade ? Madame la ministre, les maires sont habitués à gérer et à évaluer les situations d'urgence. Si l'un d'entre eux appelle au secours, c'est que la situation est grave ! Ma question est la suivante : au regard des changements climatiques, pensez-vous revoir les critères de classement en zone de catastrophe naturelle

en cas de dégâts provoqués par une tempête. Je tiens d'abord à vous confirmer les informations qui vous ont été communiquées par les services de la préfecture de l'Aube. Les dégâts provoqués par le vent sur des biens assurables entrent dans le champ de la garantie catastrophe naturelle seulement lorsqu'il a présenté les vitesses et caractéristiques fixées par le code des assurances, c'est-à-dire lorsque les vents maximaux

les particuliers et les entreprises sinistrés victimes des vents violents seront indemnisés dans le cadre de leur assurance, sans qu'il soit besoin qu'intervienne au préalable une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les effets des vents violents sont couverts

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues,

Cette loi substitue au critère classique du domicile fiscal celui de la nationalité : tout Américain doit déclarer et payer des impôts aux États-Unis. Il s'agit là d'un bouleversement considérable de la législation fiscale américaine. Le FATCA affecte en particulier les « Américains accidentels ». Il s'agit de nos compatriotes nés aux États-Unis à l'occasion d'un bref séjour, d'une escale ou visite touristique ou d'une hospitalisation.

En 2014, ils ont découvert qu'ils devaient avoir des relations suivies avec les États-Unis en matières fiscale et bancaire. En effet, leurs banques françaises les ont informés cette année-là de l'existence du FATCA. Ils devaient, dès lors, payer leurs impôts aux États-Unis. Ils ont appris que le FATCA était d'application rétroactive sur plusieurs années, avec des indemnités et pénalités de retard à la clef

Ils étaient donc tenus de remplir les formulaires envoyés par leurs banques, pour transmission au fisc américain. Ils devaient avant toute chose obtenir un numéro de sécurité sociale américain, démarche complexe pour nombre d'entre eux, beaucoup ne parlant même pas anglais. Je souhaiterais vous lire quelques extraits d'un témoignage reçu récemment : « Je suis née aux USA, en Californie, à Pasadena, de parents tous les deux Français. [ ...] Mes parents sont rentrés en France lorsque j'avais 16 mois. [ ...] « En juin 2016, ma banque m'a envoyé un courrier m'indiquant que je présentais " un indice d'américanité Je travaillais alors à plein temps et je rédigeais une thèse pour une formation que j'avais décidé de suivre pour ma carrière professionnelle. [ ...] « J'ai entrepris les démarches difficiles pour collecter les informations nécessaires à la constitution du dossier pour obtenir le numéro de sécurité sociale américain. J'ai interrompu tous mes projets personnels. [ ...] J'ai appris début 2018 que le fisc français avait transmis mes soldes bancaires au fisc américain. « J'ai engagé un cabinet spécialiste de la fiscalité française et américaine pour des honoraires estimés entre 13 000 et 15 000 euros suivant un taux horaire non contrôlable. [ ...] Le cabinet m'a indiqué que je dois en outre payer 25 000 euros au fisc américain. [ ...] « J'espère que la procédure sera terminée fin juin 2018 car, dans le cas inverse, le préjudice financier sera encore plus important puisque la France passe au prélèvement à la source et, de ce fait, je n'aurai aucun crédit d'impôt à déduire des impôts que je devrai aux USA en 2018. » Voilà une femme de cinquante-trois ans qui voit partir en fumée tous ses rêves et ses économies Les banques françaises sont en effet tenues de faire le signalement de leurs clients américains et de transmettre au fisc américain quantité d'informations. Nos compatriotes jugent cette démarche très intrusive et considèrent qu'elle porte atteinte à leur vie privée. La loi FATCA a prévu des sanctions fort dissuasives. Pour les banques, il s'agit d'une retenue à la source punitive de 30 % sur l'ensemble des flux financiers versés depuis les États-Unis sur des comptes de, voire le retrait de la licence bancaire aux États-Unis. Aucune banque ne peut donc se permettre de refuser l'application du FATCA. Quant aux « Américains accidentels », ils s'exposent à des poursuites du fisc américain, qui peut demander au fisc français d'engager des poursuites contre eux. Ils doivent également éviter de voyager aux États-Unis, sous peine de devoir y rester ... jusqu'à ce qu'ils aient régularisé leur situation. En France, les « Américains accidentels » rencontrent de grandes difficultés auprès des banques et des sociétés de gestion de portefeuille, soumises aux contrôles stricts de l'autorité américaine de régulation des marchés. Soucieuses de ne pas devenir les proies de contrôles intrusifs du fisc et de l'autorité américaine de régulation des marchés, les banques et les sociétés de gestion de portefeuille françaises sont de plus en plus réticentes à conserver une clientèle d'« Américains accidentels La plupart des banques françaises refusent l'ouverture de comptes à ces personnes, les privant ainsi de tous les services bancaires, tels que prêts, produits d'épargne retraite, cartes bancaires, etc. Elles peuvent même unilatéralement décider de fermer les comptes de leurs clients habituels dont elles apprennent qu'ils présentent un « indice d'américanité en cas de refus d'ouverture d'un compte bancaire, le code monétaire et financier prévoit une procédure de recours auprès de la Banque de France, qui peut enjoindre à une banque d'ouvrir un compte à Comment ne pas s'interroger aussi sur la légalité du « fichage » des « Américains accidentels » au regard de la loi Informatique et libertés, en raison des conséquences dramatiques qui peuvent en résulter ? J'ai, en ce qui me concerne, commencé à travailler sur ce sujet dès juin 2015, après m'être entretenue avec l'une de ces victimes résidant à Singapour. J'ai alors adressé un courrier à M. Michel Sapin, en septembre 2015, auquel a répondu M. Jean-Marc Ayrault en juillet 2016. Je vous Le fondement de l'impôt sur la nationalité et non sur le domicile fiscal relève de la compétence souveraine des États-Unis, sur laquelle la France ne peut intervenir Plusieurs « Américains accidentels » ont donc décidé de renoncer à la nationalité américaine, mais on a du mal à imaginer la complexité et surtout le coût de cette procédure. Il faut prendre un avocat américain si l'on veut que la procédure aboutisse. On m'a signalé des honoraires oscillant entre 10 000 et 100 000 euros. Une famille a dû se défaire de tout son patrimoine immobilier en France. Il faut aussi acquitter une taxe de 2 500 euros auprès de l'administration américaine et surtout, évidemment, s'être mis en règle avec le fisc américain, après avoir payé les arriérés d'impôts, les pénalités de retard et les amendes De plus, on vient de m'informer que le Congrès américain a voté en décembre 2017, il y a donc moins de cinq mois, une nouvelle loi qui aggrave considérablement la situation des « Américains accidentels »

Quelle est la finalité de cette proposition de résolution ? Agir à un triple niveau. Au plan international, l'Association des « Américains accidentels », dont je salue les efforts, a saisi le président Trump. Notre excellent collègue Antoine Lefèvre, président du groupe d'amitié France-États-Unis du Sénat, avec lequel je me suis entretenue avant son départ pour accompagner la visite d'État du président Macron à Washington, a immédiatement agi auprès des autorités américaines au plus haut niveau. L'Association des « Américains accidentels » souhaite une remise en cause de l'accord franco-américain de 2013. Elle souligne que les États-Unis ne respectent pas la réciprocité en matière d'échange d'informations entre l'administration américaine et le fisc français, ce qui pourrait nous permettre de dénoncer cet accord. Elle demande la prise de dispositions transitoires pour le passé, et l'ouverture de la possibilité de renoncer à la citoyenneté américaine selon une procédure simplifiée. le président de l'Association des « Américains accidentels », Fabien Lehagre, a saisi le Parlement européen d'une pétition transmise à la commission des pétitions, qui a déclaré la demande recevable. Elle prépare une proposition de résolution, qui sera examinée en séance plénière du Parlement européen en juin. Une résolution du Parlement européen apporterait un grand appui à cette juste cause, en mobilisant la Commission européenne sur le sujet. Au plan national, plusieurs d'entre nous ont multiplié les démarches auprès des gouvernements successifs. À plusieurs reprises, M. Jean-Marc Ayrault m'a indiqué qu'il comprenait les difficultés des « Américains accidentels », en renvoyant à des discussions entre notre ambassade et les autorités américaines. J'ai déposé cette proposition de résolution, cosignée par une centaine de mes collègues, eux-mêmes saisis de ce problème dans leurs circonscriptions. Je les remercie de l'intérêt qu'ils ont porté à cette situation. L'Assemblée nationale a repris le flambeau en créant une mission d'information sur la situation des Français nés aux États-Unis au regard du FATCA, dont les deux rapporteurs sont MM. Marc Le Fur et M. Laurent Saint-Martin. Elle m'a auditionnée le 18 avril dernier. la CNIL, a été saisie par un particulier de la question de la fermeture des comptes à partir d'un fichage des. Enfin, l'Association des « Américains accidentels » a formé devant le Conseil d'État un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 25 juillet 2017, qui constitue l'une des modalités de mise en oeuvre de l'accord franco-américain d'application du FATCA. En agissant de concert à ces trois niveaux- bilatéral, européen et national-, je suis persuadée que nous pourrons avancer vers la solution qu'espèrent nos compatriotes « Américains accidentels C'est une question de justice. Nous ne pouvons pas permettre que ces compatriotes soient pris en otages et aient à payer une rançon pour avoir le droit de vivre dignement. Je vous remercie par avance de votre soutien

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est en ma qualité de président du groupe d'amitié France-États-Unis du Sénat que je prends la parole sur cette proposition de résolution relative à la situation des « Américains accidentels concernés par le FATCA, que j'ai volontiers cosignée. Notre collègue Jacky Deromedi s'est saisie avec énergie de ce dossier. C'est un vrai sujet que celui de ces « Américains accidentels », nés sur le territoire des États-Unis mais n'y ayant séjourné que quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours, et considérés, du fait du droit du sol, comme Américains. Les voilà depuis quatre ans, du fait de l'application du fameux FATCA adopté à Washington en 2010 et en vertu d'un accord bilatéral de 2014, destinataires de courriers de leurs banques leur demandant de communiquer leur numéro d'identification fiscale américain ou d'apporter la preuve qu'ils ont renoncé à la nationalité décident de manière unilatérale de fermer leurs comptes bancaires. Les États-Unis sont le seul pays au monde à faire reposer la taxation sur la citoyenneté plutôt que sur le lieu de résidence : c'est la. Les « Américains accidentels » sont aujourd'hui contraints de rentrer dans le système fiscal américain avant de pouvoir éventuellement en sortir. Notre collègue Jacky Deromedi a explicitement décrit les affres fiscales qui découlent du FATCA pour les particuliers : en vertu d'une convention bilatérale, les impôts payés en France par les ressortissants américains ne viennent en effet qu'en déduction des taxes

Enfin, cela ne dispense pas de devoir faire des déclarations rétroactives sur les trois, voire les six, dernières années et de payer l'éventuel surplus. De plus, quelques banques profitent de la situation pour pousser dehors leurs clients présentant cette fameuse « américanité » et les traitent comme des parias.

et le représentant Mark Meadows a présenté un projet de loi complémentaire à la Chambre américaine, en vue de corriger les effets pervers de l'extraterritorialité de la législation américaine. Or, en novembre, selon l'un des défenseurs, « il n'y avait rien dans le texte de la Chambre des représentants ni dans celui voté par la commission des finances du Sénat qui aide les Américains expatriés ou les Américains accidentels Ceux-ci, qui comptaient donc sur la réforme fiscale du président Trump, ont subi une forte déconvenue. Parallèlement, en France, l'Association des « Américains accidentels », créée en 2015 et animée par son dynamique président Fabien Lehagre, a engagé une procédure devant le Conseil d'État pour s'opposer à l'application en France du FATCA, au motif que ; « aujourd'hui, l'accord n'est pas mis en oeuvre de façon réciproque par les États-Unis. Or un accord international ne peut être appliqué en droit interne qu'à condition qu'il le soit de façon réciproque. » À l'Assemblée nationale, la mission Le Fur-Saint-Martin de la commission des finances instruit ce dossier et vérifiera, en particulier, si nos banques n'interpréteraient pas à l'excès les demandes des États-Unis.

J'ai aussi pu rencontrer le président du du Congrès, le sénateur du Delaware Christopher Coons, avec qui nous avons échangé sur ce sujet. Nos collègues parlementaires américains sont bien conscients des difficultés engendrées par le FATCA.

dans cette nasse. En conclusion, je voudrais vous livrer les paroles d'un chef d'entreprise dont la banque va clôturer, unilatéralement, les comptes des différentes sociétés sociétés : « Et quelle tristesse que de voir mon pays, jadis tellement libre et courageux, capable autrefois de sortir de l'OTAN pour garder sa liberté de parole et de décision, ce pays de tout temps à l'avant-garde dans la défense sincère des plus belles valeurs humaines, quelle tristesse, donc, que de voir ce même pays se soumettre aujourd'hui, et supporter que certains de ses résidents se voient interdire, par une autre nation, de devenir entrepreneurs ou de solliciter un crédit immobilier. » Mes chers collègues, il apparaît important de soutenir la demande d'un traitement dérogatoire pour les « Américains accidentels » leur permettant soit de renoncer à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite,

Les Français ayant le statut de résident fiscal aux États-Unis peuvent ainsi se retrouver dans l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire en France. En outre, les personnes

que nous examinons vise à encourager le Gouvernement à poursuivre son action diplomatique en vue d'obtenir la réciprocité dans la mise en oeuvre de l'accord bilatéral relatif au FATCA et de permettre aux « Américains accidentels » d'être exonérés de ces obligations fiscales américaines.

Nous soutiendrons ce texte pour les recommandations qu'il avance. Effectivement, il conviendrait d'assortir d'un amendement particulier l'accord bilatéral entre la France et les États-Unis. Notre diplomatie, dans le cas présent, se doit d'agir de manière urgente et volontariste pour qu'une législation américaine appropriée soit mise au point, afin d'obtenir un traitement dérogatoire pour les « Américains accidentels », qui leur permettrait soit de renoncer à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite, soit d'être exonérés des obligations fiscales aux États-Unis. L'action diplomatique est aussi nécessaire pour que les engagements de réciprocité intégrale pris par l'administration américaine dans le cadre de l'accord dit « FATCA » soient tenus. Cette réciprocité est effectivement car, il convient de le rappeler à ce stade, dans l'accord de 2014 les États-Unis s'étaient engagés à fournir à la France des informations sur leurs ressortissants évadés fiscaux aux États-Unis. Or, à ce jour, les États-Unis n'ont engagé aucune démarche pour assurer ces échanges d'informations.

Cette arme de lutte contre l'évasion fiscale a été créée par l'administration américaine en 2010 et mise en place à partir de 2014. Que dit cette loi ? Elle fait obligation aux banques du monde entier de communiquer au Trésor américain les noms de leurs clients américains détenant plus de 50 000 dollars chez elles, sous peine, cela a été rappelé, de s'exposer à de lourdes sanctions en cas de non-coopération. Cela peut prendre la forme d'une amende équivalant à 30 % des revenus produits aux États-Unis, voire à l'interdiction pure et simple d'activité sur le sol américain par retrait de licence ou d'agrément. des mesures drastiques, dont il m'appartient de rappeler ici qu'elles devraient s'appliquer aussi aux cinquante entreprises américaines qui auraient stocké, selon la presse, 1 600 milliards d'euros dans des paradis fiscaux. Voilà un vrai cas d'évasion fiscale ! L'ONG Tax Justice Network, dans son rapport annuel publié en janvier dernier, classait les dix premiers paradis fiscaux mondiaux selon leur indice « d'opacité ». La Suisse venait en tête, suivie de très près par les États-Unis, dont l'ambivalence sur le sujet est confirmée par l'existence de ces trois États américains en situation de « paradis fiscal » que sont le Delaware, le Wyoming et le Nevada. On y autorise en effet avec une grande facilité l'enregistrement d'entreprises prête-noms et de trusts anonymes dans la plus grande discrétion ... Les États-Unis combattent l'évasion fiscale qui nuit à leurs intérêts propres. La puissance de l'économie américaine donne aux États-Unis la capacité d'imposer des règles en dehors de leurs frontières, et cela vaut aussi pour les banques du monde entier, qui doivent respecter la loi nord-américaine, puisqu'aucune d'entre elles ne pourrait se permettre de se passer de ce marché. La piste de la renégociation de la convention fiscale franco-américaine peut aussi être envisagée, mais cette procédure risquerait à l'évidence de prendre plusieurs années. Aussi, les recommandations portées par la proposition de résolution nous semblent constituer pour l'heure la voie la plus raisonnable à suivre. C'est donc ce qui nous amènera en toute lucidité à émettre un vote favorable sur cette proposition de résolution présentée par notre collègue Jacky Deromedi. La parole est à M.

de nombreuses demandes d'inscription. Elle compte bien sûr beaucoup de Bretons. Je tiens d'ailleurs à saluer son président Fabien Lehagre, qui est présent aujourd'hui, car c'est en partie grâce à lui, à son dynamisme et à la médiatisation de son action que nous avons connaissance

chers collègues, nous sommes réunis pour débattre de la proposition de résolution déposée par notre collègue Jacky Deromedi, qui a pour objet le sort de certains de nos concitoyens, mieux connus désormais sous le nom d'« d'« Américains accidentels », aujourd'hui placés dans l'obligation légale de répondre aux injonctions du fisc américain. Rappelons que cette situation est la conséquence de la loi FATCA, en vigueur depuis le 1 juillet 2014, qui oblige par effet de ricochet tous les citoyens français ayant un « indice d'américanité »- j'ai été, comme Richard Yung, surpris par ces termes-à régulariser leur situation auprès de l'administration fiscale américaine.

que l'on pourrait tout autant qualifier d'ubuesque. En effet, ces citoyens, qui sont des personnes ordinaires, vivent, travaillent, paient leurs impôts et sont en règle avec les lois de leur pays de résidence, la France. Or l'application de la loi FATCA met ces citoyens français, « Américains accidentels », dans une situation intenable,

personnes victimes- le mot n'est pas excessif -d'un détournement du droit. Nos concitoyens concernés peuvent en théorie abandonner leur nationalité américaine, mais cette renonciation ne peut être obtenue sans la régularisation au préalable de leur situation fiscale sur le territoire américain. Or ce processus étant long, complexe et, de surcroît, coûteux, les personnes touchées par l'application de cette loi sont dans l'incapacité de se charger seules de la démarche et doivent donc recourir à une aide juridique.

Certes, plusieurs scandales de fraude fiscale- nous connaissons tous ceux de la banque UBS en 2008 et, plus récemment, des « Panama papers » ou des « Paradise papers » -légitiment l'échange automatique de données entre les États. Chacun ici en est persuadé. Toutefois, dans le cas présent, il s'agit évidemment d'autre chose, et j'insiste avec force sur la nécessité de protéger les droits de nos concitoyens injustement mis en cause par l'application de cette loi. Je veux à cet égard rappeler le manque de considération des institutions fiscales américaines envers nos concitoyens. Le contraint ces derniers à payer des impôts en France et outre-Atlantique, dans la mesure où l'administration américaine, l', ou IRS, contourne l'interdiction de la double imposition, établie par la convention fiscale bilatérale du 31 août 1994, en imposant des éléments qui des éléments qui ne le sont pas en France. Il s'agit d'une unilatéralité agressive, à laquelle s'ajoute une intrusion, par l'entremise des banques, dans la vie privée de chaque citoyen franco-américain et de son conjoint, ce qui n'est pas sans poser question au regard de l'article 9 de notre code civil, d'autant plus que

que, toutes tendances confondues, les parlementaires se mobilisent sur ce sujet révélateur d'une manière très particulière de concevoir les relations internationales. Nos entreprises elles-mêmes, ainsi que les autres entreprises européennes, pourraient d'ailleurs, avec le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, se trouver confrontées à l'extraterritorialité du droit américain. Certes, on doit reconnaître l'engagement dans ce dossier du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui a porté le débat à l'échelle européenne. l'objectif demeure que cette situation trouve aussi rapidement que possible une solution définitive et ne se reproduise plus à l'avenir. C'est la raison pour laquelle la proposition formulée par notre collègue visant à entamer la négociation d'un amendement à l'accord fiscal bilatéral me semble particulièrement bienvenue. Ainsi, les négociations devraient porter sur la possibilité pour nos concitoyens de renoncer, s'ils le souhaitent, à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite- ou, à tout le moins, peu onéreuse-, mais également, pour ceux qui ne désirent pas la perte perte de leur double nationalité, la fin d'une imposition fiscale non fondée par les institutions américaines. Enfin, concernant la fermeture abusive des comptes bancaires, il est important de rappeler une nouvelle fois à nos concitoyens concernés qu'un recours auprès de la Banque de France est possible. devrait même être facilité, afin de contraindre les banques appliquant cette procédure, qui, il faut le rappeler, est contraire au droit au compte garanti par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, d'accepter la réouverture d'un compte sans usage d'une réponse dilatoire. Puisque nous en sommes à évoquer la loi FATCA, je note que cette dernière impose également aux États-Unis d'Amérique un principe de réciprocité complète. Il faudrait en bonne logique que les institutions bancaires américaines fournissent des informations à notre administration sur des comptes détenus sur le sol américain en cas d'évasion fiscale avérée. Ce principe n'étant pas respecté, une action diplomatique plus globale serait dans l'ordre des choses.

de résolution que nous examinons aujourd'hui est la conséquence de la ratification par la France, le 29 septembre 2014, de l'accord bilatéral France-États-Unis relatif à la loi FATCA, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale.

D'une part, aux États-Unis, le droit du sol est total : une personne née sur leur territoire est de fait américaine. D'autre part, seuls les États-Unis appliquent à tout Américain un impôt fédéral, quel que soit son lieu de résidence. Ces deux particularités du système américain ont conduit des Français nés accidentellement aux États-Unis à devenir des contribuables américains sans avoir de liens familiaux dans ce pays, sans y résider et même parfois sans en maîtriser la langue. Nous pouvons nous demander combien de nos compatriotes se trouvent ainsi piégés : des centaines, des milliers, sans doute, mais aucune information précise n'existe à leur sujet.

vivent sur notre territoire. Je souhaite que la Banque de France soit interrogée et qu'elle puisse nous répondre, comme elle l'a fait aux États-Unis, sur le nombre précis de personnes concernées par cette situation. En ratifiant la convention relative à la loi FATCA, l'État français a obligé nos banques à déclarer

Le syndrome de la BNP, qui a été pénalisée à hauteur de 9 milliards de dollars, a laissé une trace indélébile, qui explique la frilosité de nos apparaît clairement de reprendre les négociations par la voie diplomatique pour corriger les accords de 2014, en prenant en considération ce qui a probablement échappé aux rédacteurs de l'époque. Il me semble qu'il n'y a que deux solutions. La première consiste à laisser à nos ressortissants la possibilité de renoncer à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite. Aujourd'hui, ils doivent se plier à une démarche lourde et souvent menaçante-

La seconde solution consisterait tout simplement à ce qu'ils soient exonérés d'obligations fiscales américaines. Cette action diplomatique doit être menée à l'échelon français, c'est vrai, mais également au niveau européen, avec l'ensemble de nos partenaires qui sont dans notre situation.

Qu'en est-il des autres États européens ? Comment réagissent les établissements bancaires des autres pays ? Pouvez-vous nous éclairer sur ces sujets ? La première conséquence de cet abus du droit américain est la crainte des institutions financières françaises. Celles-ci redoutent de ne pas respecter à la lettre des engagements de la France vis-à-vis des États-Unis relatifs à la communication de leurs données clientèle. Elles craignent de devoir supporter de lourdes sanctions, de voir leur réputation entachée, voire d'être bloquées dans leur activité aux États-Unis. Sans pour autant approuver cette position, on peut comprendre dans ces conditions, mes chers collègues, que certaines banques préfèrent fermer ou refuser l'ouverture des comptes des « Américains accidentels », plutôt que d'avoir à assumer des risques liés à une ratification dont elles ne sont pas à l'origine. Notre rôle, celui du politique, des parlementaires, du Gouvernement, est de briser cet engrenage qui contraint nos banques et pèse sur nos concitoyens. Bien des interrogations restent en suspens, notamment quant au nombre de personnes concernées- je l'ai dit-, aux contraintes qui pèsent sur les banques françaises- jusqu'où doivent-elles aller ? -, à la situation des autres ressortissants européens nés aux États-Unis, à la réaction des autres États à travers le monde, au comportement des établissements bancaires dans d'autres pays, aux conséquences imposées par les États-Unis en cas de retrait de nationalité, aux conditions de la réciprocité, aux effets induits pour les membres de la famille de ces Américains dits « accidentels », puisque certains peuvent être inquiétés, aux héritages, aux contrôles, à la suspicion, etc. Toutes ces questions mériteraient un travail approfondi, qui serait qui serait bien mené s'il était confié à une mission sénatoriale, afin d'identifier des solutions politiques structurelles et durables à la problématique de l'application du droit fiscal américain sur notre territoire, sujet beaucoup plus global qu'il serait bon de traiter au fond et dans le détail.

Même si, en France, nous sommes attachés à une imposition à raison de la résidence, et non de la nationalité, nous ne pouvons que prendre acte des décisions fiscales américaines. En revanche, il nous revient de défendre les droits de nos ressortissants. Plus de 10 000 Français seraient concernés, souvent nés sur le sol américain pendant l'expatriation de leurs parents, mais n'ayant conservé aucune attache dans ce pays, certains ne connaissant même pas leur situation. Nous sommes très nombreux à avoir reçu des témoignages décrivant leur situation ubuesque. Il faut absolument que l'État français agisse pour que ces ressortissants puissent renoncer à leur nationalité américaine. Pour cela, il faut négocier une procédure dérogatoire, simple et gratuite. Aujourd'hui, renoncer à la nationalité américaine coûte, cela a été dit, très cher : il faut régulariser sa situation fiscale sur cinq ans, payer une taxe importante correspondant à la clôture des frais de dossier et régler des frais d'avocat élevés du fait de la complexité de la procédure. Cette démarche porte également atteinte à la vie privée : il faut fournir une multitude de renseignements, notamment sur ses études, ses employeurs, son état civil. Ces exigences sont inacceptables pour des Français n'étant américains que par accident, j'allais dire presque par hasard. Par ailleurs, nous devons garantir à ces « Américains accidentels » le droit au compte bancaire. Tous nos ressortissants, y compris lorsqu'ils vivent à l'étranger, ont le droit de détenir un compte bancaire en France. Ce principe- je le rappelle-avait été inscrit dans la loi à la suite de l'adoption de l'un de mes amendements en 2011. Il est anormal que des banques françaises, par peur des autorités américaines ou par volonté d'éviter les complications engendrées par la loi FATCA, puissent décider de fermer un compte en banque uniquement sur des « indices d'américanité La liberté contractuelle ne doit pas aller à l'encontre des droits humains les plus basiques. En effet, sans compte en banque, comment vivre et opérer aujourd'hui ?

Une convention fiscale permet, en principe, d'éviter les cas de double imposition : un impôt réglé dans un pays étranger est déclaré dans le pays de résidence où il permet de bénéficier d'une déduction. Avec les États-Unis, la base de taxation a évolué de manière très différente. Certaines cotisations privées pour la retraite ou la vente de la résidence principale, déductibles en France, sont imposables aux États-Unis. De même, la CSG française n'est pas considérée comme un impôt par les États-Unis et n'est donc pas déductible dans ce pays. Ainsi, s'agissant de la convention fiscale, l'enjeu dépasse de loin les seuls « Américains accidentels », mais concerne tous nos compatriotes établis aux États-Unis. Une action diplomatique résolue auprès de nos partenaires américains était plus qu'urgente. Je remercie mon collègue Antoine Lefèvre de son action à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Je remercie également très vivement ma collègue Jacky Deromedi d'avoir été à l'initiative de cette proposition de résolution, ainsi que nos collègues députés, qui se sont également saisis de ce sujet par une proposition de résolution. Je leur souhaite un plein succès, puisque Marc Le Fur et Laurent Saint-Martin se sont vus confier une mission dont nous attendons avec impatience les résultats. En effet, ce sujet, je le répète, est d'une grande importance et d'une grande urgence.

et de l'accord conclu entre Washington et Paris, un an plus tôt, pour qu'il soit appliqué sur le territoire français, les banques se trouvent contraintes d'identifier et de déclarer auprès de l'administration américaine les clients présentant des « indices d'américanité Les banques doivent depuis lors analyser un certain nombre de pièces et de documents fournis par le client avant de fournir les informations détaillées des comptes concernés à l'agence du gouvernement fédéral américain chargée de collecter l'impôt et de veiller au respect des lois fiscales encadrant le budget fédéral américain. Dans ce contexte, le principe de la fiscalité fondée sur la citoyenneté conduit à ce que soit considérée comme contribuable américain toute personne détenant la nationalité américaine, alors même qu'elle résiderait à l'étranger. Dès lors, dans le cadre de la législation actuelle, nombreux sont nos concitoyens ayant acquis la nationalité américaine à la naissance, à l'occasion d'une résidence occasionnelle ou d'un voyage de leurs parents par exemple, sans pour autant avoir résidé aux États-Unis. À cet égard, nombre d'entre eux n'ont bien souvent pour seul lien avec ce pays que celui de la naissance. Depuis l'entrée en vigueur en 2013 de l'accord conclu entre la France et les États-Unis et en 2014

En effet, abusivement considérés comme « résidents fiscaux américains », ces Français, « Américains accidentels », se sont vus réclamer des sommes importantes par l'administration fiscale américaine, alors qu'ils n'ont, dans la majorité des cas, jamais travaillé ou vécu aux États-Unis. Au surplus, ce processus de mise en conformité fiscale ou de renonciation à la citoyenneté américaine se révèle extrêmement onéreux et compliqué. En effet, les Français « américains accidentels » se trouvent contraints de payer une indemnisation correspondant à la clôture de leurs frais de dossiers. À cela s'ajoutent encore les frais d'avocats nécessaires à la régularisation de leur situation. la renonciation à la citoyenneté américaine suppose une régularisation de leur situation fiscale auprès du fisc américain sur une période de cinq ans, puis le paiement d'une taxe.

le droit au compte bancaire pour les « Américains accidentels ». Il recommandait par ailleurs d'informer les Français vivant aux États-Unis des conséquences fiscales liées à leur expatriation et de garantir la réciprocité dans la mise en oeuvre de l'accord bilatéral FATCA. Richard

Au début de 2016, les commissions des affaires étrangères et des finances de l'Assemblée nationale décidaient conjointement de constituer une mission commune d'information sur l'extraterritorialité de certaines lois américaines. Cette mission commune

d'une disposition législative américaine, que les Américains accidentels puissent renoncer à la nationalité américaine par une procédure simple et gratuite ou être exonérés de leurs obligations fiscales américaines. Enfin, la mission appelait le Gouvernement à exercer l'action diplomatique nécessaire pour que soient tenus les engagements de réciprocité pris par l'administration américaine dans le cadre de l'accord FATCA. Ces différentes recommandations n'ont, pour l'heure, pas été suivies d'effets. La proposition de résolution de notre collègue Jacky Deromedi s'inscrit dans la continuité de ces différentes initiatives et de ces recommandations. Elle vise à assurer, dans un premier temps, le droit au compte bancaire des « Américains accidentels ». Elle préconise en outre que soit garantie la réciprocité dans la mise en oeuvre de l'accord bilatéral relatif au FATCA. Elle prévoit aussi la meilleure information des Français

D'ailleurs, quand cet accord entre la France et les États-Unis a été ratifié, le 29 septembre 2014, l'étude d'impact annexée au projet de loi de ratification évoquait très rapidement cette situation, sans en mesurer toutes les conséquences.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui résonne fortement avec l'actualité internationale, marquée par le rejet récent, par le président des États-Unis, de l'accord sur le nucléaire iranien. d'un exemple supplémentaire des conséquences négatives de l'unilatéralisme américain, qui se manifeste dans de nombreux domaines : sanctions économiques contre des entreprises françaises à l'étranger, rejet de l'accord de Paris sur le climat, et, maintenant, loi FATCA, qui, malgré des intentions louables, s'est transformée en enfer administratif et fiscal pour certains de nos concitoyens. Tandis que, en France, le droit du sol est soumis à certaines conditions de résidence, les États-Unis appliquent un droit du sol inconditionnel ; toute personne née sur le sol américain possède la nationalité américaine, sans condition de résidence, même si ses parents sont étrangers. Ainsi, une personne née sur le sol américain, mais n'y résidant pas, voire n'y ayant jamais résidé, est considérée par les autorités américaines comme une personne américaine, une « ». Depuis l'adoption, en 2010, de la loi FATCA, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale des citoyens américains et contre le blanchiment d'argent, tout établissement bancaire dans le monde doit identifier les clients présentant des « indices d'américanité » et déclarer leurs avoirs à l', l'IRS, le fisc américain. En cas de manquement à cette loi, la banque doit s'acquitter d'une retenue à la source de 30 %, cela a été dit. Toutefois, les informations à fournir vont au-delà des simples informations fiscales ces « Américains accidentels » doivent fournir de nombreuses informations personnelles, ainsi que celles de leur conjoint, même si celui-ci n'a pas la nationalité américaine. Au total, on considère que plusieurs dizaines de milliers de citoyens français sont concernées. C'est par l'accord bilatéral de 2013-2014 que la France a accepté ces conditions ; c'est peut-être notre tort ... Si les autorités américaines doivent également transmettre des informations sur les citoyens français résidant sur le sol américain, en pratique, l'accord est très asymétrique, et les États-Unis reçoivent un ensemble d'informations bien plus large que ce qu'ils transmettent. Dans le rapport de juillet 2014 de la commission des finances du Sénat relatif à la loi de ratification la réciprocité était considérée comme une « question centrale ». Pour régulariser leur situation auprès des autorités américaines, les « » n'ont d'autre solution que de régler des impôts aux États-Unis ou de renoncer officiellement à la nationalité américaine.

En octobre 2016, les députés Karine Berger et Pierre Lellouche ont publié un rapport d'information sur l'extraterritorialité des lois américaines. Ce rapport montre comment le caractère incontournable du marché américain et de ses dispositions législatives permet aux États-Unis d'imposer leurs règles aux autres États. D'ailleurs, cette extraterritorialité ne concerne pas que les « Américains accidentels », puisqu'elle s'applique aussi aux citoyens américains expatriés, qui doivent déclarer leurs revenus à l'IRS. en droit américain, l'impôt est prélevé sur le fondement de la citoyenneté et non sur celui de la seule résidence- cela pourrait être amené à changer avec la réforme fiscale en cours outre-Atlantique. Dans le contexte de mobilisation croissante en France, en Europe et dans le monde, la résolution proposée par notre collègue Jacky Deromedi semble bienvenue. Elle reprend des recommandations du rapport de Karine Berger et de Pierre Lellouche et elle incite le Gouvernement à reprendre les négociations avec les autorités américaines, afin d'amender l'accord bilatéral de 2013 ou de modifier la loi FATCA pour tenir compte de la situation des « Américains accidentels secrétaire d'État, elle invite le Gouvernement à agir auprès des États-Unis pour faire respecter les engagements de réciprocité. Enfin, elle demande d'assurer l'accès normal aux services bancaires pour les particuliers touchés par la loi FATCA, de mieux informer les Français résidant aux États-Unis des conséquences fiscales de leur expatriation, pour eux et éventuellement pour leurs enfants qui naîtront sur le sol américain.

il est difficilement tolérable qu'elles menacent des familles entières de clore leurs comptes pourtant ouverts il y a des dizaines d'années. J'ai été le témoin, lors d'une permanence dans le département dont je suis élue, de la détresse de plusieurs personnes, qui en viennent à redouter toute démarche bancaire par crainte d'une transmission de leurs données à l'IRS, qui ne peuvent pas solliciter de tutelle sur le compte de leurs parents vieillissants,

C'est le résultat de plusieurs dispositifs, dont l'effet cumulatif a bien été rappelé. Tout d'abord, en matière de fiscalité, chaque pays est souverain et les États-Unis connaissent le principe de l'imposition sur le fondement de la citoyenneté. Or celle-ci peut s'acquérir par la seule naissance sur le sol américain, cela a été dit. Des citoyens français, qui ont aussi la nationalité américaine, sont ainsi tenus par le droit américain de procéder à une déclaration de

occasion-, visait à lutter contre l'évasion fiscale, un objectif qui n'est pas contestable en soi, mais qui, on le voit, a des effets pervers. Cet accord fixait un cadre pour l'échange automatique d'informations fiscales permettant de garantir une sécurité juridique des institutions financières françaises. Il faut aussi

doubles nationaux souhaitant accéder à certains produits financiers des justificatifs qui attestaient de la régularité de leur situation auprès des services fiscaux américains. Pour certains de nos compatriotes qui possèdent également la nationalité américaine du fait de leur naissance sur le sol américain, l'impact de ce dispositif a pu devenir un casse-tête administratif et financier. En l'absence de lien substantiel avec les États-Unis, pays dans lequel ils ne résident pas la plupart du temps, ils rencontrent des difficultés pour fournir les informations exigées par les établissements financiers français, notamment un numéro d'identification fiscale américain. Conscients de ces difficultés, nous avons exploré avec le ministère des finances différentes pistes, qui recoupent

Le premier enjeu a consisté à clarifier le statut des « Américains accidentels » et à fournir à ces derniers des informations utiles pour faciliter leurs démarches. À notre demande, l'ambassade des États-Unis à Paris diffuse désormais sur son site internet

préoccupations. Quelques semaines plus tard, les services fiscaux américains- l'ou IRS-avaient accordé un assouplissement des procédures relatives à la transmission par les banques des numéros d'identification fiscale des particuliers. Mais, là encore, nous devons aller plus

Toute l'équipe, qui est devant vous, se prépare donc à prendre l'avion et à aller négocier pied à pied avec nos homologues américains

plusieurs aménagements possibles, pour que les citoyens français concernés puissent bénéficier d'une obtention et d'une transmission simplifiée du numéro d'identification fiscale américain ou TIN. Nous souhaitons que les « Américains accidentels » puissent

est close. Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. Mes chers collègues, je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote.